J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020,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

La première est assez simple : nous nous trompons de cible. La deuxième est que cette taxe pourrait induire des effets pervers de report vers la consommation d'alcools plus forts. Troisièmement, nos viticulteurs et producteurs d'alcool n'ont pas été consultés.

alors, adopter une taxe sur les boissons peu alcoolisées ? Cette taxe pourrait avoir un effet négatif induit, celui de reporter la consommation de ce type de boissons peu alcoolisées, qui titrent à moins de 10 degrés, vers des alcools plus forts. Cet article est par ailleurs un très mauvais signal

%, ce qui compte pour nous, c'est vraiment le message de santé publique envoyé à une jeunesse qui démarre en général sa consommation alcoolique ces produits extrêmement sucrés, avec un impact à la fois sur l'entrée dans l'alcoolisation et sur l'obésité- cela a été dit hier.

afin de décourager l'entrée précoce des jeunes dans la consommation d'alcool par le biais de boissons très sucrées masquant la présence et le goût de l'alcool. deux, en 2004, par la loi relative à la santé publique, cette taxe est désormais de 11 euros par décilitre d'alcool pur. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, cette taxe a eu pour effet de limiter le marché français des premix : moins de 10 000 litres en ont été vendus en 1997, contre 950 000 litres en 1996, alors que ce marché était en plein essor. Selon une étude du même observatoire, la nouvelle hausse intervenue en 2004 a conduit à une chute de 40 % des ventes de premix en 2005. Pourtant, certains industriels de l'alcool ont exploité une faille de la loi de 2004, qui excluait les vins aromatisés du champ d'application de la taxe. C'est ainsi que l'on a vu apparaître des vins ou cidres aromatisés, ciblant clairement les jeunes par un emballage, un marketing ou une appellation, et offrant des prix bas auxquels les jeunes sont particulièrement sensibles. Ainsi, selon le propriétaire de la marque Rosé Sucette, « ces bouteilles, à moins de 3 euros sur linéaire, seront un tremplin permettant aux néophytes d'accéder aux vins plus classiques. Notamment pour un public plutôt jeune et féminin Il s'agit là d'une porte d'entrée clairement identifiée vers l'alcoolisation des jeunes. Le présent amendement vise dès lors à étendre aux boissons aromatisées à base de vin

les boissons alcoolisées spécifiquement tournées vers l'alcoolisation des jeunes- c'est bien clair. Certaines boissons, du fait de leur composition

pour cibler les populations les plus fragiles, en particulier les jeunes, mais aussi- j'y reviendrai peut-être tout à l'heure -les femmes enceintes, dont la consommation d'alcool peut

L'éducation et la prévention doivent être privilégiées- cela a été dit -plutôt que de s'orienter vers de nouvelles taxations, qui ne sauraient résoudre les problèmes d'addiction ou de consommation à risque. Réaffirmons l'existence d'un modèle de consommation responsable conciliant art de vivre et préservation de la santé de nos concitoyens.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

à tenir compte d'une réalité : contrairement à ce que vous dites, madame la ministre, ou à ce que dit M. le rapporteur général, aucune étude d'impact n'a été faite sur les conséquences pour la viticulture française de l'instauration de cette taxe.

J'ai le plus grand respect pour celles et ceux qui sont tentés de défendre des intérêts économiques ; naturellement, ça compte ! Cela dit, la lutte la lutte contre le développement de l'alcoolisme chez les jeunes, et même chez les plus jeunes, me semble un objectif de santé publique majeur. Or, mes chers collègues, pour lutter contre l'addiction au tabac, je ne compte ni sur Philip Morris ni sur Marlboro

celui de l'implication de la filière dans la prévention en direction des femmes enceintes. Sans aide, sans financement public- personne ne l'a salué, j'aimerais au moins pouvoir le dire au nom de la filière -, nous avons investi, nous tous, viticulteurs, 100 000 euros. Il était de

qui englobe la totalité des problématiques de l'alcoolisation au travers des effets de cette taxe.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Je suis impliquée dans la vie publique depuis maintenant vingt ans. Je suis passée par tous les arcanes du mandat local maire adjointe de la première ville de Martinique, qui compte près de 100 000 habitants, conseillère générale d'un canton de 17 000 habitants 100 % populaire, conseillère régionale, première vice-présidente de la région en charge des politiques publiques importantes, et depuis deux ans sénatrice, sans compter une bonne vingtaine d'années d'action militante pure.

qu'ils ont à l'époque tenus sous tutelle, je réponds que je suis parfaitement majeure et que je sais de quoi je parle

L'an dernier, à la même époque, la décision a été prise d'augmenter de manière extrêmement importante la taxe sur le rhum, sous des prétextes de santé.

Il est vrai que le jour où il a prononcé ce discours et quitté le pays, nous subissions sur le tarmac de l'aéroport un violent tremblement de terre ; c'était peut-être un signe. Quel est l'avis de la commission ? commission ? Nous avons adopté l'an dernier à une large majorité un alignement très progressif, madame Conconne, de la fiscalité sur les spiritueux dans les DOM sur celle qui est applicable en France Cet alignement, qui ne débute qu'à partir du 1 janvier 2020, s'effectuera jusqu'en 2025, ce qui laisse tout de même largement le temps à la filière de s'adapter.

pour cette fois. Les alcools forts sont en moyenne beaucoup plus consommés que dans l'Hexagone, c'est un fait. Le baromètre de Santé publique France a d'ailleurs fait apparaître, en 2014, que les DOM se plaçaient au sein des régions les plus concernées par la consommation d'alcool à risque de dépendance, dont font partie, bien sûr, les spiritueux. En outre, le syndrome d'alcoolisation foetale fait

vote. Il n'est pas question de stigmatiser un alcool plutôt qu'un autre. Le syndrome d'alcoolisation foetale, mon confrère Jomier l'a rappelé, touche tous les alcools. Toutefois, les alcools forts, et le rhum en fait partie, ont des effets toxiques plus importants, et c'est une réalité.

Je ne peux pas partager ce point de vue. Pour moi, la Martinique, qui est un producteur d'alcool comme bien d'autres départements de France, fait partie du territoire français et, pour reprendre l'expression d'Olivier Dussopt, la France est une et indivisible. Le terme de « néocolonialisme » au

des bouleversements importants auraient été engagés dans les politiques publiques. Ce n'est pas le cas chez moi ! Ce n'est pas le cas en Guadeloupe ! Ce n'est pas le cas à La Réunion, qui chauffe régulièrement ! Voilà pourquoi je dis que je ne suis pas la France ! C'est scandaleux

Ce n'est pas les uns contre les autres. Ce n'est pas un département contre un autre. C'est la France dans sa globalité, métropole et outre-mer

Mes chers collègues, je vous appelle au calme et vous invite à respecter les orateurs qui s'expriment et à modérer vos propos. Je souhaite que nos débats conservent la sérénité qui fait la marque de fabrique de la Haute Assemblée et contribue à la bonne image de nos travaux. En tout état de cause, je n'hésiterai pas, afin de maintenir la sérénité de nos débats, à faire usage des prérogatives que le règlement confère à la présidence de séance. Je vous rappelle ainsi de l'article 33, alinéa 4, de notre règlement : « Si les circonstances l'exigent, le président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. » L'article 93, alinéa 2, dispose pour sa part : « Est rappelé à l'ordre tout orateur qui s'en écarte et tout membre qui trouble l'ordre

Je prends la parole pour apaiser un peu les débats. Chacun a ses arguments. Chacun s'exprime avec sa force de caractère et sa personnalité.

de la Guadeloupe ou des départements producteurs de rhum ne sont pas moins attentifs que nous à la lutte contre l'alcoolisme. Je crois même qu'ils doivent l'être encore plus, au

Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les onze degrés. En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d'alcool, jusqu'à seize degrés ou dix-sept degrés, dont la cible principale est la jeunesse, même si celle-ci Dans une démarche de prévention, l'objet de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique, afin de dissuader les plus jeunes de les acheter. Pour l'heure, en effet, il n'y a aucune distinction d'un point de vue fiscal entre les bières à six degrés et les bières à seize degrés. cet amendement s'appuient sur une recommandation de la Ligue contre le cancer et de l'Institut national du cancer, qui rappellent que l'alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France. Enfin, il convient de préciser que, selon les catégories d'alcools et de boissons alcoolisées, les taux des droits qui leur sont appliqués varient également et sont tout aussi importants. À ce jour, si les vins dits « tranquilles » sont taxés à hauteur de 3,82 euros par hectolitre, d'autres demeurent, quant à eux, plus importants. C'est notamment le cas des vins mousseux, 9,44 euros par hectolitre, mais aussi des vins doux naturels, 47,67 euros par hectolitre, dont le taux d'alcool commence à partir de quinze degrés.

ne sont généralement pas proposées par la grande distribution. Les dispositions de cet amendement s'appuient sur une recommandation de l'Institut national du cancer, qui rappelle que l'alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France.

titrant généralement à 8,5 % et parfois jusqu'à 10 %, voire 12 %, soit autant que des vins. Ces bières ont un succès important, notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité. Or une canette de cinquante centilitres d'une bière titrant 8,5 % ou plus représente trois à quatre unités d'alcool. Outre la quantité d'alcool, le conditionnement, en particulier la canette en métal, pose problème, dans la mesure où celle-ci ne peut pas être refermée. Cela incite à terminer chaque canette entamée, avant de se rendre dans un lieu où l'usage d'alcool est interdit ou impossible- je pense par exemple au milieu scolaire ou professionnel, aux lieux d'accueil, d'accueil, aux administrations ou aux enceintes sportives -ou de commencer une activité. Il en résulte une alcoolisation importante et rapide, avec un pic d'alcoolémie atteint au bout de trente minutes, qui augmente le risque d'effets dommageables pour la personne : accidents de la route, violences, risques socioprofessionnels, comportements à risque, etc. L'objet du présent amendement est de limiter la consommation de ces produits par l'extension d'une taxe sur les bières titrant à 8,5 % et plus. Actuellement, elle existe déjà pour les bières de plus de 18 %. Les jeunes ayant globalement un plus faible pouvoir d'achat que la population générale, ils sont très sensibles à l'effet prix, comme vient de le démontrer l'Écosse, avec l'instauration d'un prix minimum. Il s'agit ainsi de limiter le caractère incitatif à l'achat et donc à l'alcoolisation excessive,

et la volonté du Gouvernement de mieux prévenir les risques liés à la consommation excessive d'alcool, laquelle constitue la deuxième cause de cancer évitable. En effet, l'offre de bières fortes titrant généralement à 8,5 %, voire à 12 % ou à 16 %, se développe de plus en plus : 12 %, c'est autant que le vin. Or ces boissons fortes connaissent un certain succès, notamment auprès des publics jeunes. C'est d'autant plus regrettable que ces bières sont souvent distribuées dans des contenants d'un demi-litre et contiennent, de fait, une grande quantité d'alcool. d'exemple, une canette de 50 centilitres d'une bière à 8,5 % représente 3,5 unités d'alcool, soit près de deux fois la quantité maximale journalière recommandée par la médecine.

Merci, madame la ministre, pour vos explications. Je connais votre implication dans le domaine de la prévention. Je retire cet amendement, qui est un amendement d'appel. J'ai conscience qu'il faut laisser le temps aux filières de revoir le conditionnement en canettes. Ce sera là une preuve de leur implication dans la prévention et dans la lutte contre la consommation excessive d'alcool des jeunes.

à tous ceux qui le souhaitent, et uniquement à eux, de s'inscrire dans cette démarche, de tester leur addiction, parfois sous forme ludique, parfois sous forme de défi personnel. Le Gouvernement ne franchit pas ne franchit pas le pas qui sépare la prévention de la prohibition. Il n'y aura pas de campagne de prohibition ou de mise sous séquestre de je ne sais quelles bouteilles. Nous laissons les acteurs de la prévention mettre en place les initiatives qui sont les leurs. Pour notre part, nous en restons à la politique de prévention qui est la nôtre.

1613 telle qu'elle avait été conçue dans la loi du 30 décembre 2017. La réduction de la consommation de sucres, notamment de boissons sucrées, constitue un enjeu majeur de santé publique, largement reconnu sur le plan scientifique. Dans son rapport de décembre 2016, rappelle que « la contribution des sucres à l'excès d'apport énergétique ne doit pas être négligée, notamment pour le diabète de type 2, le cancer de l'endomètre et le cancer du sein la santé (OMS) a appelé à réduire l'apport en sucres dans la ration énergétique journalière à 10 %, soit environ 200 kilocalories. Le réduire à 5 %, soit 25 grammes de sucre par jour, abaisserait le risque de surpoids, d'obésité et de carie.

commission ? Monsieur Bonhomme, je comprends parfaitement vos arguments, mais il me paraît prématuré de relever les tarifs de la taxe

ce phénomène en 1997 au titre des grandes épidémies. C'est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l'origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. au-delà du prix humain et social qu'elles font supporter aux patients, représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise donc à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop élevée. Le produit de cette taxe serait affecté à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette taxe comportementale viendrait compléter la démarche d'éducation à la santé et la politique de prévention mise en oeuvre par le ministère de la santé à travers la généralisation du Nutri-score- à défaut d'avoir

elles seules favoriser la survenue du cancer. Il semble donc plus prudent d'attendre les conclusions des enquêtes conduites par les agences sanitaires afin d'évaluer l'opportunité d'une nouvelle taxe alimentaire

Cette disposition est entrée en vigueur le 1 juillet 2018. S'il convient de saluer l'impact relatif de cette modulation, force est de constater que certains industriels contournent toutefois encore cette nouvelle taxe en diminuant la contenance de leurs bouteilles, tout en augmentant leur prix.

Quel est l'avis de la commission ?